Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en demandant l'organisation de ce débat, la délégation aux entreprises a voulu se faire l'écho des centaines d'entrepreneurs qu'elle a rencontrés depuis sa création. création. Depuis deux ans, nous sillonnons le territoire ; partout, le poids de l'administratif est vécu par les entreprises comme l'un des premiers blocages à leur développement. Ce blocage se décline en excès de normes, en maquis de règles, en rigidité, en instabilité : plus les entreprises se voient imposer de règles, plus leur espace de liberté est réduit, ce qui nuit à leur créativité et à leur croissance.

Selon le critère du poids de la réglementation, la France est classée 115 sur 138 pays par le Forum économique mondial. C'est une piètre performance ! Il s'agit donc d'un enjeu économique majeur, car notre compétitivité et notre attractivité De nombreux pays européens l'ont bien compris et se sont saisis du problème. On peut se demander si la France a bien pris la mesure de l'enjeu, même si le Président de la République a annoncé en mars 2013 un « choc de simplification ». Qu'en est-il quatre ans plus tard ? La délégation aux entreprises s'est saisie de cette question en adoptant le rapport, qu'elle avait confié à Olivier Cadic et à moi-même. Pour élaborer ce rapport, nous avons effectué des déplacements en Europe afin de comprendre la démarche de simplification menée par plusieurs de nos voisins : l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas. Nous avons ensuite entendu à Paris une vingtaine d'acteurs qui sont au coeur du sujet : d'abord, les représentants des entreprises et de ceux qui les accompagnent pour gérer la complexité ; ensuite, les institutions chargées de la simplification, à commencer par le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, M. Jean-Vincent Placé, qui aurait dû être présent aujourd'hui. Comment interpréter sa défection, Vous nous direz si nous devons y voir un désintérêt pour le sujet, ce que je n'espère pas, ou, peut-être, l'expression d'une difficulté à assumer un bilan délicat ... Nous avons également entendu des acteurs extérieurs au Gouvernement, mais bien placés pour analyser la situation française, que ce soit à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes ou chez France stratégie. Enfin, nous avons exploré certaines idées avec les membres de et des universitaires. La volonté de simplification, affichée en haut lieu, a-t-elle produit des résultats pour les entreprises françaises ? L'inflation législative ne date pas d'hier, mais, fait nouveau, elle va en s'accélérant. Si le nombre de projets de loi évolue peu, leur volume augmente, notamment à la faveur de leur examen au Parlement : le nombre d'articles des projets de loi est en moyenne doublé à l'issue de la navette. On a tôt fait d'accuser les parlementaires, mais le Gouvernement est comptable du cinquième de cette dérive imputée aux amendements. En outre, pour légiférer, le Gouvernement recourt à l'ordonnance aussi bien qu'au projet de loi, contribuant ainsi directement à l'hyperactivité législative, sans l'aide du Parlement. S'ensuit mécaniquement un emballement réglementaire, toutes ces normes enchevêtrées créant de la complexité et de l'insécurité juridique. L'Union des industries chimiques nous a transmis une courbe frappante qui manifeste l'emballement normatif depuis une quinzaine d'années, ne concerne-t-elle que le domaine de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Il aurait été intéressant d'avoir la même courbe en matière fiscale ou de droit du travail. La France resserre encore un peu plus cet étau normatif en transposant souvent les directives européennes au-delà des obligations standards, ce qui disqualifie nos entreprises et, même, les incite à délocaliser leur production. Cela fait des années que l'on tente d'améliorer la situation sans grand succès visible, malgré le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, un secrétaire d'État dédié, un conseil de la simplification pour les entreprises et un gouvernement qui se félicite d'avoir initié 463 mesures de simplification. Toutefois, l'élan initial s'est rapidement essoufflé. Le 10 juin 2015, M. Thierry Mandon annonçait, pour le 1 juillet 2015, la mise en place d'un comité permettant d'expertiser les études d'impact du Gouvernement.

carrément usurpée, voire à effet ... Tout cela forme un tableau pointilliste : la politique de simplification n'arrive pas à convaincre, prise entre effets d'annonce et difficultés de mise en oeuvre. D'ailleurs, 43 % des mesures annoncées par le Conseil de la simplification ne sont pas effectives. On évoquera des blocages, qui tiennent à la résistance au changement de ceux à qui profite la complexité, mais il faut aussi reconnaître que la volonté politique du Gouvernement a été défaillante. Pourtant, le Gouvernement soutient que son action a dégagé une économie potentielle pour les entreprises d'environ 5 milliards d'euros annuels. Un tel chiffrage, effectué à partir des études d'impact produites par l'administration, reste invérifiable. Aucun audit préalable n'a été fait. Surtout, il néglige le coût qui résulte du flux parallèle d'obligations nouvelles : pénibilité, compte personnel de formation, transition énergétique ... Si les entreprises ne ressentent pas un choc de simplification, elles ressentent assurément un choc de réglementation Or il est tout à fait possible de réussir : nos voisins d'Europe du Nord, eux, ont misé durablement sur l'amélioration de leur réglementation. L'Union européenne elle-même s'est engagée dans une telle démarche : sous l'impulsion du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le flux de textes nouveaux a objectivement ralenti. Que conclure de nos déplacements en Europe ? Là où elle fonctionne, la simplification est un objectif politique, généralement transpartisan, qui mobilise l'ensemble du Gouvernement. L'évaluation préalable des coûts y est perçue comme un moyen de rendre efficace la décision politique, pas de s'y substituer. La simplification obéit à une méthodologie rigoureuse et repose sur des objectifs et le suivi d'indicateurs. Surtout, des résultats chiffrés et vérifiés sont obtenus. L'Allemagne a ainsi allégé le coût de la bureaucratie pour ses entreprises de 14 milliards d'euros entre 2006 et 2011. Enfin, la réduction du stock de règles s'articule souvent avec une régulation du flux de normes, grâce à une règle de compensation entre création et suppression de normes. Dans tous ces pays, un organe indépendant contrôle la qualité des études d'impact, sur lesquelles repose le pilotage de la simplification pour les entreprises. Chacun de ces organes est doté d'un collège de quelques membres experts issus du monde économique, sans mandat politique ni fonction administrative. Il rend un avis qui est publié en même temps que le texte du projet de loi ou de règlement envisagé. La majorité sénatoriale s'est également saisie du sujet et a présenté de nombreuses propositions. Des mesures d'ordre général, comme le, ou la fin de la surtransposition des normes européennes. Nous avons également fait adopter au Sénat des mesures attendues par les entreprises, malheureusement balayées d'un revers de main par le Gouvernement

; Jean-Baptiste Lemoyne y reviendra certainement. Je laisse maintenant le soin à Olivier Cadic de présenter la suite du rapport de la délégation : il analysera la situation française, au regard des enseignements que nous avons pu tirer de nos observations à l'étranger,

Tel Ulysse, notre délégation propose une odyssée en quatre étapes pour simplifier la vie des entreprises et augmenter notre efficacité. À l'étranger, la simplification est un processus méthodique. Chez nous, elle tient plutôt du mirage politique. C'est le fameux « choc de simplification », qui a eu trois visages en trois ans.

La simplification, c'est un instrument de compétitivité qui doit s'imposer aux politiques sectorielles. Or les ministères continuent à élaborer des normes indépendamment les uns des autres, et à en rajouter par rapport aux règles européennes sans se soucier de l'impact économique global. Bref, les acteurs de la simplification s'épuisent en vidant la mer avec une cuillère.

Le principe semble acquis, mais les ordonnances, les propositions de loi et les amendements y échappent encore. Surtout, l'exercice reste trop formel pour être utile : ces études d'impact sont de qualité inégale et sont souvent réalisées au dernier moment. Le Parlement ne s'en est donc pas emparé. Et le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel, le Secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'État n'a pas permis d'en améliorer la qualité, si bien que notre pays continue à légiférer pour un oui, pour un non, avec entrain, ce qui rend fous les entrepreneurs ! Quant à l'évaluation rétrospective des lois, elle est loin d'être systématique. Même si tout n'est évidemment pas chiffrable, il n'y a que la comparaison dans le temps et dans l'espace qui permette de mesurer l'écart produit par une réglementation publique. Dans ce contexte, annoncer la suppression d'une norme pour toute norme nouvelle, la fin des surtranspositions de textes européens et la généralisation des tests PME sans appliquer ces mesures ne peut que créer de la désillusion. Pour s'attaquer à la simplification, la France traite le symptôme plutôt que le mal. Nous devons assumer notre responsabilité collective et nous interroger sur nos méthodes, sans quoi le fardeau administratif des entreprises ne pourra pas être allégé. Nous proposons donc quatre étapes dans l'odyssée qui nous mènera à bon port. consiste à penser la simplification comme un processus qualité. Quelle entreprise peut fonctionner sans service qualité ? Ce n'est pas un hasard si certaines entreprises réussissent alors que d'autres disparaissent. Nous devons créer ce service qualité pour la règle de droit. Sous la houlette du Premier ministre, un réseau dédié au sein du Gouvernement mobilisera tous les ministères sur cette question pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Sa première mission sera de chiffrer la charge administrative supportée par les entreprises : il s'agit de savoir où nous en sommes et de pouvoir nous comparer avec nos voisins. On nous oppose que ce chiffrage coûterait 3 millions d'euros. Qu'est-ce par rapport aux gains substantiels que nous pouvons attendre de cette méthode qui a fait ses preuves chez nos voisins ? Nous pourrons ensuite arrêter des objectifs de réduction nette de la charge bureaucratique- comme l'a fait l'Allemagne, à hauteur de 25 % en quatre ans -, des indicateurs et des règles pour y parvenir. L'établissement d'un plan de réformes globales, au début de chaque mandat, évitera que les dispositions juridiques applicables aux entreprises soient modifiées plus d'une fois par législature. Leur impact sera étudié en amont, leurs objectifs seront chiffrés et les indicateurs à suivre définis : l'étude d'impact deviendra ainsi l'outil principal de qualité de la norme. Une clause de révision devra aussi être insérée dans chaque loi pour évaluer son efficacité dans les cinq ans suivant son adoption. Ainsi, l'élaboration des lois obéira à un processus d'amélioration continue. La roue de Deming décrit ce cercle vertueux : préparer, exécuter, contrôler, ajuster. deuxième étape consiste à alléger le stock normatif. Nous avons deux siècles de lois derrière nous : pour commencer, il faut élaguer le stock de normes et l'alléger des règles devenues obsolètes avant d'en créer de nouvelles. La collaboration déjà engagée entre entreprises et administration doit se poursuivre il faut réévaluer la nécessité des règles et procédures qui compliquent la vie des entreprises. L'objectif est de parvenir à des simplifications substantielles. Ce travail doit mieux être articulé avec l'échelon européen, à la fois avec Bruxelles et avec les autres États européens. Nous devons comparer la performance de notre réglementation avec celle d'États voisins qui partagent des exigences comparables aux nôtres, en termes de santé publique, de protection du consommateur et de sécurité industrielle. Les salariés français sont-ils en meilleure santé que leurs voisins grâce à l'existence d'une médecine du travail ? Nos raffineries pétrolières sont-elles plus sûres grâce à une législation plus stricte ? Non : les raffineries françaises concourent pour 26 % des accidents en Europe alors qu'elles ne représentent que 10 % des sites. L'efficacité des règles juridiques doit s'apprécier à l'aune de résultats concrets. consiste à concevoir la régulation au service des entreprises. Pourquoi faire porter la responsabilité à un fonctionnaire de déterminer ce qui est autorisé ou pas ? Passons d'un système où tout est interdit sauf ce qui est autorisé à un système où tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ainsi nous libérerons non seulement les entreprises, mais aussi l'administration. La régulation doit se faire par objectif et non par moyen. Plus libre, l'entreprise sera plus responsable. Il convient aussi de porter à l'échelon européen nos exigences nationales. La transposition de directive doit se faire de manière stricte. Si, ensuite, nous voulons poser des exigences supplémentaires, cela doit faire l'objet d'un texte distinct, dont l'impact devra être évalué. Enfin, notre pays doit cesser d'anticiper sur les règles européennes à venir. La quatrième étape consiste à mieux légiférer. Le Parlement est comme une usine à produire des lois. Seul un processus qualité pour leur élaboration peut garantir leur efficacité et leur simplicité. En amont, il faut associer les entreprises à l'élaboration des lois : acceptons de prendre ce temps-là, car il est déterminant pour améliorer non seulement la qualité, mais aussi la légitimité, et donc l'effectivité de la loi. La réalisation d'un test PME sur les projets de textes qui leur sont applicables doit devenir obligatoire. Faciliter les expérimentations en amont est aussi un moyen de mieux calibrer les règles avant leur adoption. Nous devons également miser sur l'étude d'impact préalable, qui doit être approfondie, et poser d'abord la question de l'utilité d'une nouvelle règle. également obligatoire pour les projets d'ordonnances et les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour. Surtout, sa qualité doit être contrôlée par le Conseil de la simplification pour les entreprises, dont nous proposons de transformer les missions et la composition pour en assurer l'indépendance. Le Conseil rendrait un avis consultatif, mais public sur l'étude d'impact, afin de créer du débat public et de l'émulation entre ministères. Enfin, au Parlement, la procédure d'examen des textes pourrait être améliorée. Nous suggérons un débat d'orientation préalable avant d'attaquer l'examen d'un projet de loi concernant les entreprises. Nous proposons de réfléchir à de nouveaux outils pour endiguer le gonflement des textes au cours de la navette. Nous voulons qu'un nouveau regard soit porté sur l'activité des parlementaires, un regard qui ne se réduise pas à mesurer combien de textes ou d'amendements ils déposent. Nous demandons une mise à jour de l'étude d'impact après la première lecture. Enfin, nous voulons développer une culture d'évaluation préalable au Parlement. Le contrôle de l'efficacité des lois adoptées doit également être renforcé. Leur déclinaison réglementaire doit mieux respecter la volonté du législateur. Voici l'essentiel de nos propositions pour simplifier efficacement et libérer nos entreprises. Il s'agit de revoir en profondeur nos façons de faire, au bénéfice de la compétitivité de nos entreprises. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent », aurait dit Albert Einstein.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 28 mars 2013, le Président de la République lançait le programme dit du « choc de simplification », censé rendre plus lisibles et plus rapides les normes et les procédures administratives pour les citoyens et les entreprises. Un premier projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives fut voté le 20 décembre 2014. Le sujet n'est pas mineur pour notre pays. Un Français sur quatre estime ses relations avec l'administration complexes. Pis, selon le, le classement international de la France en termes de fardeau administratif s'est dégradé au fil des années pour atteindre la 121 place en 2015. Du point de vue des entreprises, les contraintes administratives sont une réalité bien connue. Démarches longues, procédures complexes, multiplicité des interlocuteurs, renseignements inadaptés à des situations particulières, manque de réactivité des services sont des phénomènes qui pèsent particulièrement sur nos PME et nos TPE. Pourtant une simplification de 25 % des charges ferait économiser 15 milliards d'euros aux entreprises, dégagerait des gains de productivité et,, contribuerait à soutenir la croissance et à libérer l'emploi. Les Français ne demandent qu'à entreprendre librement et à prendre des initiatives, comme l'a montré le succès du statut d'auto-entrepreneur, mais ils ne pourront le faire que dans un cadre administratif favorable susceptible de comprendre et de répondre à leurs attentes. La loi du 20 décembre 2014 a mis en place un certain nombre de mesures allant dans le bon sens, mais largement insuffisantes. Elles sont mises en place pour la première fois par un secrétariat d'État dédié explicitement à la simplification depuis juin 2014. Ont été ainsi votées, entre autres mesures, la réduction du nombre de commissions locales compétentes en matière d'aménagement du territoire et de services au public, la suppression ou la simplification des régimes d'autorisation préalable et de déclaration pesant sur les entreprises ; la simplification du code du commerce la transposition de deux directives sur les marchés publics ; la suppression d'obligation de déclaration pour la participation au développement de la formation professionnelle. Au regard de l'immensité de la tâche de simplification à accomplir, au niveau tant local que national, cette loi paraît bien timide. Il faut d'ailleurs noter qu'en février 2016 seulement 56 % des mesures à destination des entreprises étaient effectives. Lors du déplacement de la délégation sénatoriale aux entreprises, dont je suis membre, dans mon département des Hautes-Alpes le 30 juin 2016, avec sa présidente Élisabeth Lamure et nos trois collègues Michel Canevet, Guy-Dominique Kennel et Michel Vaspart, la rencontre avec les entreprises et les acteurs de terrain avait permis de mesurer que la complexité et, surtout, l'instabilité normative sont des griefs récurrents faits à l'État. constat lors de chacun de nos déplacements. Un an et demi après le vote de la loi, l'édiction permanente de nouvelles normes, notamment sur l'accessibilité, l'environnement ou les enseignes, réduit les marges et empêche la création d'emplois. Un dirigeant d'une PME locale ironisait également sur le fait qu'il aurait besoin d'un équivalent temps plein administratif uniquement pour s'adapter aux mises à jour normatives de notre législation Il apparaît enfin que l'inadéquation de notre réglementation à la réalité des PME reste un problème majeur. Le cadre réglementaire de l'accès aux marchés publics s'avère particulièrement difficile à appréhender. Les règles de rédaction écartent de fait nombre de PME par manque de compétences. La réglementation est bien souvent inadaptée au caractère saisonnier de l'économie locale. On pourrait évoquer aussi le manque d'interlocuteurs fiables capables d'aider des entreprises, qui ont le sentiment d'être livrées à elles-mêmes dans les abysses administratifs. Si le « choc de simplification » a certes permis quelques avancées, elles sont systématiquement remises en cause par les législations et des contraintes supplémentaires. Dans les Hautes-Alpes comme dans les autres départements, le compte pénibilité et le futur prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sont des sources d'inquiétudes pour nos entrepreneurs, car ces mesures sont non seulement difficiles à mettre en place, mais aussi très coûteuses. Et ce ne sont pas seulement les entrepreneurs qui sont victimes de ce trop-plein normatif ! Ce sont d'abord les employés, dont les salaires pourraient augmenter si leurs entreprises ne subissaient pas un tel fardeau. On assiste en réalité au mouvement suivant : un pas de simplification en avant, deux pas de complexité en arrière. Le principal problème en France reste le volume de la législation, auquel le Gouvernement n'a jamais osé s'attaquer : 400 000 normes, 10 500 lois, 127 000 décrets Et les parlementaires que nous sommes n'y sont pas étrangers ! Ces textes sont-ils tous nécessaires ? Au Royaume-Uni ou en Italie, par exemple, l'édiction d'une nouvelle norme doit obligatoirement passer par la suppression d'une autre. La France devrait s'inspirer de ce système. Chaque loi votée devrait comporter un volet « simplification ». La fin de la surtransposition du droit communautaire, déjà prolifique en matière normative, relève également du bon sens. Le numérique permet une rapidité d'exécution et une réduction des coûts impossibles auparavant. Par exemple, pourrait être mise en place une déclaration fiscale unique et dématérialisée regroupant les impôts, la TVA, la formation continue, les déclarations de cotisation que la déclaration sur les dividendes et intérêts. En matière de droit du travail aussi la simplification tarde à aboutir. Permettre le référendum d'entreprise, instaurer une instance représentative unique fusionnant les comités sorte que les accords collectifs s'imposent effectivement au contrat de travail, instaurer la présomption de licéité de l'accord collectif sont autant de mesures qui simplifieraient réellement les relations des entreprises avec les administrations et libéreraient les énergies. L'administration, quant à elle, doit se recentrer sur les rescrits en matière de droit du travail pour une meilleure adaptation aux réalités de terrain. Pour toutes ces raisons, il est indispensable pour l'économie française que nous allions beaucoup plus loin dans la simplification

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la simplification de la vie des entreprises est une question récurrente de cette législature. Déclinée au gré des débats- simplification des normes agricoles, simplification administrative, création du Conseil d'évaluation des normes -, la simplification comme une incantation résoudrait à elle seule tous les maux dont souffre notre économie. Le débat de ce matin n'échappe pas à cette règle, puisqu'il faudrait, selon ses initiateurs, alléger le fardeau administratif des entreprises pour améliorer la compétitivité de celles-ci,

cette liste n'est-elle pas exhaustive. Pour faire moins de normes, faisons plus de normes, en somme ! Or cette inflation normative, n'est pas due qu'au zèle des administrations de l'État. Cette vision caricaturale minimise l'impératif constitutionnel de clarté du droit. Il n'y a pas de volonté perverse de quelques administrateurs, mais l'exigence de produire la la norme la meilleure au service de la sécurité juridique, voire, parfois, de corriger des erreurs du Parlement. De plus, si la norme peut être contraignante à l'égard de certains, il faut rappeler que, à plus long terme, elle en protège d'autres : c'est le cas chef du droit du travail, mais aussi des procédures administratives. Pour autant, nous ne nions pas les difficultés rencontrées quotidiennement par nos entreprises. Seulement, cette exacerbation est en grande partie liée

de nombreux services ne permet pas une prise de décision administrative dans les deux mois. On peut le regretter, mais ce sont bien les politiques d'austérité qui ne permettent pas d'évolutions significatives en la matière.

qu'une simplification du code du travail contribuerait au développement de l'activité de leur entreprise, et ils sont seulement 8 % à penser que la simplification des procédures administratives pourrait retentir sur leur activité. revanche, l'inquiétude face à l'accès au crédit reste très vivace chez les entrepreneurs. Ainsi, pour de nombreuses PME, les solutions de financement proposées par les banques demeurent

européenne, ainsi que des critères de crédit aux entreprises, lequel devrait être réorienté vers l'investissement utile, avec des taux d'intérêt d'autant plus bas que le crédit serait destiné à l'emploi, aux salaires et à la formation. Il faudrait aussi encadrer véritablement la sous-traitance, comme en Allemagne, et étendre la responsabilité des entreprises donneuses d'ordres. De même, il est indispensable de mieux contrôler les circuits d'aide publique.

Enfin, il faut renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Une des raisons des difficultés que rencontrent de nombreuses PME est la faiblesse de la demande intérieure : chômage, précarité, bas salaires, tous ces phénomènes minent la demande salariale, tandis que les politiques d'austérité budgétaire dépriment la demande publique. vous l'aurez compris, si nous souscrivons à certains éléments de l'état des lieux dressé par Mme Lamure, comme la complexification du droit, la multiplication de textes législatifs sans réelle cohérence et la pratique contestable des ordonnances, nous n'approuvons pas toutes les propositions de la délégation sénatoriale aux entreprises. Si la coproduction législative avec les entreprises peut être une piste, il ne faut pas oublier que l'État est le garant de l'intérêt général et de l'indépendance à

On le voit, ce débat n'est pas neutre politiquement. Il aura été utile, tout au moins si nous en tirons cette conséquence que l'évaluation qualitative doit l'emporter dans tous les cas sur une évaluation trop souvent faussement comptable ! La parole

Cette interrogation n'est pas nouvelle ; on en parle depuis au moins 1983 et la création d'une commission pour la simplification des formalités des entreprises. Aujourd'hui, quel est le constat ?

Une vraie méthode collaborative a vu le jour au sein d'ateliers participatifs associant les acteurs économiques et les représentants de l'administration. Composé de représentants des petites et des grandes entreprises, de parlementaires, d'experts, le Conseil de la simplification pour les entreprises s'apparente,

». Source d'une économie de 4 milliards d'euros par an pour les entreprises, ce programme se décline à travers, notamment, la déclaration sociale nominative, la DSN, les marchés publics simplifiés, la saisine de l'administration par voie électronique et le guichet Entreprises.

Nous avons tenté d'y remédier dès 2013, en créant le Conseil national d'évaluation des normes, chargé de simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

permet aux citoyens et aux acteurs économiques d'adresser des propositions au Gouvernement dans le domaine de la simplification. Il a déjà recueilli plus de 4 000 contributions et compte plus de 19 000 inscrits. 000 inscrits. Ces démarches participatives et contributives nous tiennent à coeur, à nous écologistes. Nous saluons donc les avancées de la démarche de gouvernement ouvert.

Pour ce qui est des processus de simplification concernant directement les entreprises, le site simplification. modernisation.gouv.fr en recense des domaines aussi divers que les procédures de création, les échanges avec l'administration, l'emploi, la formation et l'apprentissage, mais aussi la transmission des entreprises et les obligations comptables, sociales et fiscales.

doit permettre aux entreprises d'économiser plus de 5 milliards d'euros en 2017. Ce sera donc un gain d'attractivité et de compétitivité considérable.

qui sont des acteurs économiques essentiels. Depuis vingt ans au moins, tous les gouvernements affichent leur volonté de simplifier, selon des modalités diverses.

Par ce certificat, délivré par le préfet du département dans un délai de deux mois, l'administration s'engage à identifier les règles applicables au projet d'entreprise et à respecter un délai d'instruction pour la délivrance des autorisations nécessaires.

Les causes de ce mauvais classement sont connues et s'expliquent notamment par une instabilité réglementaire et l'insécurité juridique qui en découle, par des arbitrages gouvernementaux puis législatifs pris en l'absence d'études d'impact- il existe en effet un contournement possible de cette procédure le dépôt d'amendements, qui permet d'échapper aux contraintes constitutionnelles -et, naturellement,

Je serai plus nuancé, parce que je distingue la bonne de la mauvaise norme. La norme n'est pas mauvaise en soi, mais ses modalités d'application sont parfois kafkaïennes.

Qu'écrit M. Guérin, artisan en menuiserie dans le Morbihan ? « Je n'en peux plus des nouvelles complications administratives qui nous sont imposées sans explication et surtout sans interlocuteurs compétents et joignables !! Tout semble fait pour que toutes ces tâches administratives et juridiques ne puissent être réalisées par notre secrétaire mais confiées à des logiciels coûteux ou à des cabinets comptables qui se créent des rentes et grèvent les budgets des TPME comme la mienne

La parole est à M. Martial Bourquin, pour le groupe socialiste et républicain.

représente l'un des chantiers prioritaires de ce quinquennat. Il a pour vocation de relancer l'activité économique dans notre pays. Cette simplification administrative est largement attendue par l'ensemble des acteurs économiques et, plus particulièrement, par les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises,

et dix-huit minutes en moyenne par jour pour accomplir leurs missions quotidiennes, dont près de la moitié concernent des tâches administratives La simplification est donc un véritable enjeu pour les PME et TPE, et, plus généralement, pour l'ensemble de l'activité économique française. On sait

Il concerne l'ensemble de l'Union européenne, puisque la Commission européenne estime qu'une réduction de 25 % des charges administratives pesant sur les entreprises permettrait une augmentation de 0,8 à court terme et de 1,4 % à plus long terme. Loin de vouloir vous assommer de chiffres, je voulais simplement que l'on prenne acte de la prise en compte

Deuxième exemple, l'allégement des obligations comptables, qui s'adresse directement aux très petites entreprises. Plus de 3,7 millions de microentreprises sont concernées par la suppression de l'annexe aux comptes annuels.

que « les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations

15 000 acheteurs publics impliqués dans le développement de la simplification de l'accès des PME et TPE à la commande publique. La procédure simplifiée entraîne sans conteste un gain de temps et d'argent pour les PME et TPE. Il est également à noter que l'augmentation du seuil en dessous duquel les entreprises sont mises en concurrence est de 25 000 euros.

Votre intérêt renouvelé pour la simplification en faveur des entreprises témoigne d'un enracinement de la politique de simplification dans les moeurs administratives et politiques. C'était d'ailleurs le voeu formé par le Président de la République lors du lancement du choc de simplification, voilà maintenant près de quatre ans. Le Gouvernement a toujours conçu la simplification comme un mouvement permanent en faveur de la compétitivité de notre pays. La simplification n'est pas un élément accessoire des politiques publiques. Bien au contraire, il s'agit d'une politique structurelle qui stimule l'activité économique, en rendant les procédures plus rapides et plus aisées, sans diminuer les protections ou les droits essentiels des entreprises, des salariés ou des particuliers. À la différence de ce que certains souhaiteraient, déréguler ou porter atteinte à la santé et à la sécurité de nos concitoyens, ou encore à l'environnement. Simplifier, dans

axe est le recours à une méthode collaborative permanente : la création du Conseil de simplification pour les entreprises en janvier 2014 a associé chefs d'entreprise, élus, experts et hauts fonctionnaires. Elle a permis d'engager un travail réaliste, pragmatique, concret, de nature à simplifier la vie des entrepreneurs.

et évite de voir une bonne idée s'évanouir dans la nature, même si l'on peut toujours relever, ici ou là, telle ou telle insuffisance.

le chiffrage : il a été réalisé par un cabinet totalement indépendant du Gouvernement, et ce à la demande non pas du Gouvernement, mais du Conseil de la simplification

le rapport de votre délégation. Vous vous interrogez également, à juste titre, sur le flux des nouvelles mesures. La propension à créer de nouvelles normes, dont certaines sont parfois nécessaires,

Il serait vain de s'attaquer au stock sans oeuvrer à la réduction du flux : c'est probablement le volet le plus difficile de l'action de simplification, tant la tentation est grande de réguler ou de modifier la réglementation, pour les administrations comme pour les politiques.

Cet atelier a déjà permis des avancées significatives. Je pense notamment à la réglementation en matière d'enquête publique ou de performance énergétique. Cette méthode mérite à l'évidence d'être renforcée. Notre méthode de simplification a donné des résultats concrets : plus de 460 mesures pour les entreprises ont déjà été annoncées depuis le début du choc de simplification, outre les mesures prises à destination des particuliers et des collectivités. C'est considérable. mesures sont législatives, d'autres réglementaires, d'autres enfin découlent de simples évolutions des processus de gestion. Toutes ont été élaborées en concertation totale avec les acteurs concernés.

des marchés publics, la charte de non-rétroactivité fiscale, que nous avons signée en 2014 avec Michel Sapin et qui est respectée,

pour les entreprises important et exportant des biens, nous avons facilité les régimes dits de suspension de droits et de taxes, en supprimant toutes les formalités et cautions inutiles. J'arrête là cette énumération, pour mieux me concentrer sur un chantier emblématique auquel votre assemblée ne manquera pas d'accorder une attention toute particulière : la prise en compte des petites entreprises dans la politique de simplification. C'est un enjeu essentiel,

complexité. C'est pour cette raison que nos actions en faveur des petites entreprises se sont concentrées, en priorité, selon trois axes. En

Cette mesure concerne un million de microentreprises, de moins de dix salariés. En outre, les petites entreprises de moins de cinquante salariés ont la possibilité d'établir des états simplifiés. On estime l'économie engendrée pour les entreprises concernées à 1,1

deuxième lieu, au-delà de ces allégements importants de procédures, le Gouvernement a oeuvré à garantir une meilleure sécurité juridique, le développement du rescrit, par exemple. De la même manière, nous avons demandé à la Direction de la législation fiscale qu'elle publie ses circulaires fiscales à périodicité fixe, le premier mercredi de chaque mois, et ce afin d'éviter aux TPE et aux PME de se livrer à une veille juridique fastidieuse et coûteuse pour être informées des dernières évolutions de la réglementation. lieu, outre les mesures sectorielles que nous promouvons, un axe important de notre action en faveur des petites entreprises consiste en la facilitation des formalités d'embauche. Ainsi, nous avons pris des mesures « apprentis » permettant de lever les freins à l'embauche rencontrés par les apprentis mineurs, qui ne pouvaient être facilement recrutés

En collaboration avec les acteurs économiques, nous continuons de travailler sur des dispositions en faveur des petites entreprises, particulièrement dans le domaine de l'innovation, à travers le dispositif France Expérimentation, dont les lauréats seront présentés le mois prochain.

mais nous demeurons convaincus de son efficacité pour développer notre tissu productif, assurer le rayonnement international de nos entreprises et renforcer l'attractivité de notre territoire. Nous en